L'obligation de fourrière est une charge très lourde, notamment pour les communes de petite taille, en termes de responsabilité, d'organisation et de permanence, elle fait peser sur les communes le poids de financements très importants. L'article 3, modifié par la commission, résout la question de l'organisation des mutualisations sous forme associative, mais il nous semble indispensable, au regard de la pratique,

à alléger le texte de la commission, dans la mesure où tous ces éléments sont déjà pointés dans notre réglementation, en particulier dans l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime, par lequel les mutualisations du service de fourrière sont déjà possibles, et d'ailleurs mises en oeuvre dans bien des endroits, et où, en matière de délégation de service public, les choses sont parfaitement encadrées. Il est ainsi tout à fait possible à une association qui gère un refuge de candidater à un appel d'offres pour gérer un service de fourrière pour le compte d'une commune ou d'un regroupement,

mélanger les animaux errants issus de la rue accueillis dans des fourrières et dont le statut sanitaire est incertain avec des animaux qui sont en refuge et en attente d'être adoptés. Il était donc essentiel de lever cette confusion, qui était totalement inexplicable.

89 rectifié vise à supprimer les précisions apportées à l'Assemblée nationale et en commission au Sénat quant à la mutualisation ou à la délégation du service public de fourrière supprimer le versement libératoire introduit en commission en cas de remise directe d'un animal à son propriétaire ; à réintroduire l'alinéa relatif à la formation des gestionnaires de fourrière, avec toutefois des équivalences. Sur le premier point, la commission souhaite conserver cette nouvelle rédaction, qui consacre des modes d'organisation mis en oeuvre sur le terrain et conforte les fourrières.

Comme le souligne le rapport, la fourrière est définie comme une structure communale, un service public, qui permet l'accueil et la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais de garde. De plus, les communes peuvent déléguer le service public de fourrière à des structures privées ou associatives, plutôt que l'exercer en régie. Dans les faits, donc, de nombreuses associations se voient confier la mission de fourrière, tout en disposant, par ailleurs, d'un refuge dans le cadre de leurs activités associatives. Afin de compléter la disposition prévoyant que le gestionnaire de la structure d'accueil et de garde suive une formation en matière de bien-être des animaux de compagnie, il nous semble opportun que, dans leurs contrats de prestation, les fourrières soient tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux. La parole

monsieur le ministre,

Il est important de se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Tel est l'objet de cet amendement. La loi prévoit aujourd'hui l'identification obligatoire de la plupart des chiens et chats. Ne sont reconnus comme moyens légaux d'identification que le tatouage ou la puce électronique, certes. Notre commission n'entend pas revenir sur ce point, encadré par le droit européen. il est important d'aller vers des méthodes plus fiables et uniformes d'identification. Un animal disposant d'un collier gravé d'une adresse ne sera pas considéré comme identifié au sens de cette obligation. ailleurs, la loi précise par quels moyens la fourrière est autorisée à rechercher le propriétaire d'un animal perdu ou abandonné : le tatouage, la puce ou le collier. La rédaction de l'Assemblée nationale supprimait le collier, ce qui revenait à dire qu'une fourrière ne pourrait pas utiliser le collier d'un animal pour retrouver son propriétaire. Je considère que ce serait dommageable au bien-être animal, donc je suis défavorable à cet amendement. Quel est l'avis

que par le tatouage ou la puce électronique. Absolument pas ! Il s'agit uniquement des conditions dans lesquelles une fourrière est autorisée à restituer les animaux. Quand la rage sévissait sur le territoire national,

On le remettrait alors à la sortie du délai légal de fourrière à une association pour adoption, alors qu'il a un propriétaire, certes négligent et qui mérite peut-être d'être sanctionné pour n'avoir pas fait immatriculer son chien ? Il est hors de question d'envisager de ne pas le lui rendre. C'est simplement cela que visait

par les arrivages de chiens. C'est la raison pour laquelle, sans vouloir ajouter de la maltraitance à la maltraitance, nous avons décidé de revenir à ce délai de huit jours, qui correspond à une réalité de terrain et à une gestion plus facile pour les fourrières. Quel est

M. Arnaud Bazin. Il s'agit ici de la qualification professionnelle des salariés des élevages et des animaleries.

des chats et des lapins, par exemple, une certification professionnelle de la catégorie « chats » serait valable pour tous, y compris pour les chiens, alors que ce n'est pas le cas actuellement. Il s'agit donc d'une régression du droit existant.

En commission, sur proposition de l'auteur de cet amendement, nous avons adopté un renforcement du ciblage des qualifications professionnelles du personnel des refuges, fourrières, élevages ou animaleries. Aujourd'hui, il suffit que l'un des personnels dispose d'une qualification figurant sur une liste prévue par décret, mais non spécifique aux espèces d'animaux accueillies, en dehors des chiens et des chats. Nous avons prévu que la qualification porte sur au moins l'une des espèces accueillies. En d'autres termes, une certification relative aux poissons ne suffira pas pour un gestionnaire de fourrière de chiens et chats. À l'inverse, nous n'avons pas souhaité exiger une qualification pour chacune des espèces accueillies. Avec la diversification des animaux de compagnie, les refuges peuvent être amenés à accueillir des espèces plus diversifiées, tels que les reptiles ou les lapins. La commission a donc précisé que la qualification devait être liée à au moins l'une des espèces accueillies, toujours dans un souci de simplification. Nous ne souhaitons pas aller plus loin, au risque de pénaliser de nombreux refuges. Je souhaite rassurer le sénateur Bazin, la rédaction n'est pas moins-disante sur les chats et les

code rural et de la pêche maritime définit l'élevage de chiens ou de chats comme le fait de détenir au moins une femelle reproductrice, dont au moins un chien et un chat est cédé à titre onéreux. Il inclut donc les particuliers qui ne disposent d'aucune formation en la matière. Une visite rapide de certaines plateformes d'annonces en ligne suffit pour se rendre compte qu'il s'agit d'une pratique très répandue ; des chiens et des chats sont reproduits à domicile, avec les risques qu'une mauvaise pour la femelle qui met bas ou pour les jeunes animaux. Gérer une portée n'est pas un acte anodin et, face aux difficultés, certains propriétaires peu scrupuleux cèdent rapidement les chiots ou les chatons, alors que ceux-ci ne sont pas encore sevrés. On ne peut pas s'improviser éleveur. C'est la raison pour laquelle cette activité est réglementée lorsqu'elle s'exerce dans un cadre professionnel. Le présent amendement vise donc à étendre à tous les éleveurs de chiens et de chats, y compris aux particuliers, l'obligation d'être en possession d'un certificat ou ou d'une formation ayant permis d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie Quel est l'avis de la commission ?

Toutefois, la mesure proposée concerne ce que j'appellerais « les particuliers éleveurs », c'est-à-dire les gens comme vous et moi, dont la chienne, par exemple, a eu plus d'une portée dans l'année. Dès lors que ces animaux sont cédés, ces personnes sont considérées comme éleveurs de chiens et de chats. qu'il ne s'agit pas ici d'élevage professionnel de chiens et chats. La loi prévoit donc un régime intermédiaire : les personnes concernées doivent s'immatriculer comme éleveurs, afin d'être suivies administrativement, mais elles ne sont pas soumises aux conditions de certification, de déclaration en préfecture ou de détention des élevages professionnels. Le droit existant me semble équilibré : pour les personnes qui n'en font pas une activité professionnelle ou lucrative, mais qui vendent simplement les petits de leurs animaux de compagnie, je ne souhaite pas renforcer outre mesure les formalités applicables. Celles-ci seraient de toute façon très difficiles à contrôler et pourraient conduire à davantage d'abandons. L'avis de

aux services de la direction départementale de la protection des populations et de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Cet article, tel qu'il a été voté par les députés nous apparaît indispensable pour évaluer la situation des animaux domestiques en France et apporter des solutions pérennes visant à améliorer leur bien-être et lutter contre l'abandon. C'est la raison pour laquelle cet amendement tend à revenir sur les modifications effectuées en commission des affaires économiques restreignant ces transmissions aux carnivores et, ainsi, à assurer le suivi de l'ensemble des animaux de compagnie.

En commission, nous avons souhaité restreindre le champ des données collectées aux professionnels et associations travaillant avec les chiens et chats. Nous estimons que ces animaux sont au coeur des sujets d'abandon et, de par leur nombre en France, la priorité des politiques publiques. J'entends les arguments du Gouvernement, qui souhaite élargir à d'autres espèces le champ des données collectées,

la concertation menée avec l'ensemble des parties prenantes ne semble pas encore aboutie. Il serait dommageable de définir un texte non opérationnel sur un sujet aussi important. C'est la raison de cet amendement de suppression.

L'opposition des associations au dispositif issu de l'Assemblée nationale provenait principalement de l'exclusion des associations sans refuge du dispositif de famille d'accueil. Sur le terrain, avec les maires, ce sont près de 3 200 associations qui aident à trouver des foyers temporaires pour les animaux abandonnés, en suppléant souvent les refuges. C'est une réalité de terrain- je tiens, une fois de plus, à le souligner. Nous avons entendu ces associations, les élus et les refuges, et nous avons trouvé un point d'équilibre qui nous paraît bon. Nous avons réintroduit les associations sans refuge dans le texte, tout en leur donnant

la rapporteure. Cet amendement vise à apporter deux modifications qui satisferont une partie des points soulevés par l'amendement précédent. Il tend à corriger une erreur quant au champ des animaux pouvant être accueillis et à préciser que ce sont les membres du bureau de l'association sans refuge

dans les refuges, ces animaux proviennent soit de la fourrière au terme des délais légaux, soit d'une cession directe par leur propriétaire, soit d'une saisie à la demande de l'autorité administrative ou judiciaire. C'est ce dernier point qui manquait et qu'il me semble utile de réintroduire

93 rectifié , au profit de l'amendement n° 94 rectifié Comme je l'ai dit à l'instant, l'examen en commission a permis de considérablement enrichir cet article. Nous avons atteint un équilibre, qui me semble satisfaisant et qui a été accueilli favorablement par les associations. de M. Bazin vise à remplacer la quasi-totalité du dispositif adopté en commission par une rédaction en grande partie équivalente. Nous nous rejoignons, par exemple, sur les formalités de déclaration des associations sans refuge, la tenue d'un registre, la possibilité pour ces associations d'avoir recours à des familles d'accueil, les exigences de formation de leur personnel ou encore l'existence d'un contrat-cadre avec la famille. Sur l'ensemble de ces points, l'amendement est satisfait par le texte de la commission. Toutefois, la réécriture à laquelle il tend me paraît apporter des restrictions trop importantes au fonctionnement des familles d'accueil, en contradiction avec la souplesse que j'ai souhaité conserver.

La prolifération de chats constitue un véritable fléau et présente des risques pour leur propre bien-être, ainsi que pour la biodiversité. Or la stérilisation a un coût important, ce qui peut être rédhibitoire pour certains propriétaires, ainsi que pour les maires qui procèdent à des campagnes de stérilisation de chats errants. À des fins d'incitation et d'accompagnement, le présent amendement vise donc à appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % aux opérations de stérilisation des chats. chats. Quel est l'avis de la commission ? Enfin un sénateur qui se soucie du financement ! Cela nous fait plaisir ... Le Gouvernement demande aux maires de stériliser tous les chats de France à leurs frais. chats de France à leurs frais. La stérilisation est du ressort de la responsabilité de chacun. À l'heure où la pression fiscale est déjà forte, on ne peut faire payer les contribuables pour les propriétaires d'animaux.

rendait obligatoire la stérilisation des chats errants à la charge des collectivités. Si cette obligation a été supprimée par la commission des affaires économiques du Sénat, nous craignons qu'elle ne réapparaisse à l'occasion de la commission mixte paritaire. Les sénateurs du groupe SER comprennent parfaitement l'intérêt sanitaire et écologique de cette mesure, au sein de la Haute Assemblée, nous sommes particulièrement vigilants lorsqu'il est question de contraintes financières pesant sur les collectivités. Vous le savez, on recenserait entre 9 et 11 millions de chats errants en France en 2020. Le coût d'une stérilisation étant d'environ 70 euros pour un mâle et 130 euros pour une femelle,

que le Gouvernement s'engage, dans les trois mois à compter de la publication de la loi, à remettre un rapport au Parlement sur les dispositifs d'accompagnement financier qu'il compte mettre en oeuvre si cette stérilisation venait à devenir obligatoire. La parole est à M. Fabien Gay,

Quel est l'avis de la commission ?

également celui de l'évaluation de l'impact économique de cette opération. Les chiffres que vous avez donnés sont tout à fait exacts,

convient pas s'agissant d'un transfert de pouvoir de police et de responsabilité. En effet, les transferts obéissent à des règles strictes, prévues par le CGCT. doit par ailleurs pouvoir être rattaché à l'exercice d'une compétence communautaire, ce qui n'est pas le cas dans le texte qui nous est proposé. Cet amendement a pour objet de clarifier l'intervention de l'intercommunalité par la mutualisation de moyens- embauche de personnel, équipements dédiés, etc. -, au service des maires, et de ne pas créer une concurrence dans l'exercice des pouvoirs de police en la matière.

Le scrutin est ouvert.

Le bien-être et le comportement futur de l'animal dépend de cette période, au cours de laquelle il apprend à communiquer, à gérer son éventuelle anxiété, à contrôler les morsures ou les griffures et à s'adapter à son environnement. En cas de séparation trop précoce,

Quel est l'avis de la commission ?

L'objectif est de lutter contre les tromperies et d'éviter qu'un acquéreur ne soit encouragé à abandonner ou euthanasier les petits à naître. Pour supprimer cet article, le rapporteur a notamment argué du fait qu'il serait très difficilement applicable, faute de technique fiable de diagnostic de la gestation animale.

La suppression de cet article ne semble pas favoriser le renforcement du bien-être animal, car l'on sait le sort qui peut être réservé à des portées d'animaux non voulues.

Cependant, je ne crois pas que le niveau de trésorerie d'une personne à un instant donné soit un bon indicateur de sa capacité à prendre soin de son animal. Que le prix d'acquisition soit réglé en une fois ou en plusieurs ne permet pas non plus de distinguer les bons et les mauvais propriétaires d'animaux. J'émets donc un avis défavorable sur votre amendement.

Mon amendement ne visait absolument pas à les stigmatiser, mais uniquement à protéger chacun et à éviter des situations épouvantables, tant pour l'animal que pour les personnes,

Les grandes enseignes d'animalerie françaises ont compris l'enjeu et ne s'y opposent pas. Cette liste positive doit être édictée dans le code rural et de la pêche maritime, car elle est plus adaptée à cette réglementation. Il n'y a pas de race

qui pourront émettre un avis scientifique sur l'autorisation de détention par des personnes n'ayant pas de compétence particulière. Il est nécessaire que ceux qui seront amenés à statuer sur ce lien de connaissances

Pour mémoire, l'article 4 prévoit un basculement vers une liste positive des animaux non domestiques pouvant être détenus, dont le principe est l'interdiction de détention et les espèces listées l'exception. de l'amendement écrase la quasi-totalité des améliorations apportées en commission. Or ces évolutions sont nécessaires pour mettre le dispositif en cohérence avec le droit européen, ce à quoi nous avons travaillé. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne, qui s'est prononcée sur des listes similaires, mises en oeuvre par les pays voisins, a insisté sur la nécessité de faire preuve de souplesse et d'objectivité dans l'élaboration de la liste. La commission a ainsi apporté plusieurs compléments. Elle a instauré un comité spécialisé chargé de cette élaboration, dont la composition sera garantie par la loi. Elle a précisé les critères présidant à l'élaboration de la liste, en incluant le risque de zoonose, particulièrement pertinent en temps d'épidémie Elle a prévu une révision automatique de la liste, tous les trois ans, pour inclure ou retirer certaines espèces en fonction des avancées de la connaissance spécifique. Enfin, elle a permis aux tiers de suggérer des révisions ponctuelles de la liste. La commission ne souhaite pas renoncer à ces avancées, qui sont à la fois philosophiquement justifiées et nécessaires au respect du droit européen. En outre, nous ne souscrivons pas à l'approche proposée par l'auteur, qui prévoit que la liste n'est révisée que s'il se révèle que toute personne peut détenir l'espèce concernée, même en l'absence de connaissance préalable spécifique, sans que cela constitue un risque. Ce critère est impossible à remplir. Nul ne peut garantir le risque zéro, même dans le cas d'un chien, et pour toute personne non avertie.

En effet, il existe déjà une liste d'espèces pour lesquelles il a été estimé que la difficulté et la dangerosité liées à leur détention sont telles que celle-ci n'est autorisée que sous les conditions draconiennes fixées pour le troisième régime, à savoir l'obtention d'un certificat de capacité, doublée d'une autorisation d'ouverture.

Cela me paraît aller dans le bon sens ; plus nous sommes nombreux à oeuvrer pour la bientraitance animale, mieux nous nous portons. La commission

S'il est pertinent d'appliquer la liste positive aux particuliers éleveurs, il faut clarifier cette notion. Le renvoi au décret permettra d'ajuster les paramètres et de réaliser les consultations nécessaires. Il ne concernera que l'application du présent article, sans réinstaurer, de manière générale, une distinction entre élevage d'agrément et élevage professionnel.

Tel est l'objet de cet amendement.

sauvage protégée (I-FAP), de tous les animaux non domestiques. En effet, il n'y a pas d'intérêt à étendre les obligations d'identification et d'enregistrement à toutes les espèces animales non domestiques, car toutes ne sont pas victimes de trafic ou menacées de disparition.

En commission, sur l'initiative de notre collègue Arnaud Bazin, nous avons en effet souhaité étendre le champ d'application de l'enregistrement obligatoire des animaux non domestiques au fichier national I-FAP. Aujourd'hui, seules les espèces protégées victimes de trafic ou en disparition sont concernées. Il nous a semblé pertinent de rassembler davantage d'informations sur les spécimens détenus en France et de pouvoir mieux les relier à leurs propriétaires, que ceux-ci soient des établissements ou des particuliers qui détiennent de nouveaux animaux de compagnie exotiques. Cela permet de lutter contre l'abandon ou la perte de ces animaux mais également d'assurer un suivi des populations possédées. Toutefois, je comprends les arguments de l'auteur du présent amendement, qui estime que la généralisation totale de l'obligation d'identification est trop ambitieuse et difficile à mettre en oeuvre.

si elles ne sont pas homogènes sur le territoire et même si nous sommes convaincus que certaines animaleries font leur maximum en faveur du bien-être animal, restent insatisfaisantes dans bon nombre de cas. Les dérives qui peuvent être provoquées par la vente en animalerie ne vont pas dans le sens du renforcement du bien-être animal.

chats en animalerie, pour des raisons éthiques et sanitaires ; cette disposition ne concernerait pas les autres animaux de compagnie, tels que les lapins ou les petits rongeurs. La commission a entièrement réécrit cet article, en supprimant l'interdiction prévue et en la remplaçant par un encadrement des points de vente d'animaux, mais cela ne nous semble pas suffisant.

ailleurs, nombre de vétérinaires indiquent que les chats et les chiens issus d'animaleries souffrent fréquemment de la gale, de la teigne ou de parasites intestinaux, liés à la concentration des animaux derrière les vitrines. Or l'amendement adopté en commission ne visait à interdire que les vitrines donnant sur la rue.

Nous avons inscrit dans notre droit que l'animal est un être doué de sensibilité ; nous devons en tirer les conséquences : il ne peut constituer un produit d'appel dans une animalerie. La

l'interdiction des expositions en vitrine. Néanmoins, en dépit de toutes les précautions qui pourront être prises, la vente de chiots et de chatons en animalerie ne saurait en aucun cas être adaptée. Il est important de sensibiliser les futurs adoptants à cette question, ce qui passe par la visite de l'animal dans son environnement de départ, l'élevage, lorsqu'il est encore auprès de sa mère. Cette visite permet également de se rendre compte des conditions d'élevage et de lutter contre les trafics. Le présent amendement vise donc à interdire la vente de chiens et de chats en animalerie à compter du 1 janvier 2024 et de permettre ainsi la socialisation de ces animaux, qui commence avec la mère et l'éleveur et doit se poursuivre rapidement avec la famille d'accueil.

Je souhaite, avant toute chose, rappeler d'où nous partons sur le sujet des animaleries : l'article proposé par l'Assemblée nationale interdisait la vente de tous les animaux de compagnie : les chiens, les chats, mais également toutes les autres espèces. Je me félicite que nous revenions à un débat plus mesuré, puisque les amendements soutenus se limitent aux seuls chiens et chats. Toutefois, je n'y serai pas favorable, compte tenu des importants effets de bord de telles dispositions. Les animaleries représentent une part minoritaire des ventes en France, aujourd'hui : on parle de 100 000 animaux abandonnés par an, alors que les animaleries ne vendent que 20 000 chats et chiens chaque année. Elles ne sont donc certainement pas la seule cause de l'abandon des surtout quand on connaît leur prix de cession et quand on sait que ces animaux quittent l'animalerie vaccinés et identifiés. Au-delà de cela, ma position n'a pas changé sur le sujet. Je considère qu'il faut maintenir l'ouverture de la vente en animalerie pour deux raisons : un argument pratique et un argument juridique. En pratique, je préfère laisser exister un circuit de vente autorisé, ayant pignon sur rue, contrôlé et inspecté régulièrement par des vétérinaires, plutôt que l'interdire et fermer les yeux sur les ventes qui continueront ailleurs, hors de tout contrôle. La fermeture totale des animaleries, sans tarir la demande,

concerne l'aspect juridique, il existe une interrogation constitutionnelle : peut-on interdire à certains professionnels et certains types d'établissements uniquement de vendre des animaux, tandis que d'autres canaux équivalents seraient maintenus, sans que des critères objectifs soient cités ?

Surtout, pour inciter davantage les animaleries à se lier à des refuges ou à des fondations, comme c'est le cas en Californie, la commission a promu ces partenariats, afin que les chiens et chats qui y sont vendus puissent provenir plus souvent de refuges, ce qui est de nature à désengorger ces derniers, tout en promouvant les bonnes pratiques en animalerie. Cette position me paraît être la plus opérationnelle, car elle évite de nombreux effets de bord liés au principe d'interdiction, qui donnera immanquablement lieu à des trafics en tout genre.

Le scrutin est ouvert.

cet article est redondant. En effet, l'article L. 214-8 du code rural dispose clairement que les dispositions qu'il édicte sont applicables à toute cession effectuée par une association de protection animale. Ces cessions sont donc déjà encadrées par l'obligation de fournir un certificat vétérinaire, un document d'information, une attestation de cession, etc. Cet article est donc redondant, restrictif au-delà de l'existant

Mme la rapporteure.

en prévoyant une fermeture administrative des établissements contrevenants pour au moins deux mois. Selon un règlement européen, les mouvements commerciaux et non commerciaux d'animaux domestiques sont autorisés au sein de l'Union à deux conditions : disposer de documents d'identification valides et de la preuve d'une vaccination antirabique

Ce vaccin ne peut en effet être administré qu'à partir de douze semaines, auxquelles il faut ajouter trois semaines pour le rappel. Selon certaines animaleries peu scrupuleuses, quinze semaines, c'est encore trop- je rappelle que nous parlons d'animaux d'importation. On constate donc de nombreuses fraudes et on évoque 100 000 entrées illégales par an.

Sitôt l'infraction constatée, il n'y a plus de manquement qui justifierait, dans le droit existant, cette fermeture provisoire. C'est la raison pour laquelle cet amendement tend à prévoir la suspension automatique d'un établissement ayant commis des manquements répétés aux règles européennes sur les carnivores domestiques, chiens et chats.

contrôle de l'âge minimal d'entrée des chiots. Pour ce faire, nous avons travaillé avec un vétérinaire de la brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire.

Les agents des douanes et de l'inspection vétérinaire doivent s'assurer qu'aucun chiot d'un âge inférieur à quinze semaines n'entre sur le territoire national. Or cette non-conformité est extrêmement difficile à déterminer

Après avoir reconnu aux animaux la qualité d'êtres vivants doués de sensibilité, nous ne pouvons les vendre comme de vulgaires objets. L'utilisation de plateformes en ligne et de réseaux sociaux pour proposer des animaux de compagnie à la vente est en pleine expansion

Pour mettre un terme à ces flux, qui ne sont plus acceptables, il est essentiel d'interdire la vente d'animaux sur les plateformes et sites non spécialisés. Malheureusement, la rédaction de cet article, en évoquant les sites internet et non les plateformes, ne permet pas d'encadrer réellement cette situation. situation. Sur ces plateformes, certains vendeurs falsifient des numéros Siren pour se faire passer pour des entreprises spécialisées. La seule manière de protéger efficacement les animaux est donc d'interdire leur vente sur les sites et les plateformes non spécialisés pour permettre un contrôle plus simple et plus efficace.

Les députés ont cantonné la possibilité de cession d'un animal de compagnie sur un site internet aux personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-1

Ainsi, cet article, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, ne supprime pas la possibilité pour un particulier de proposer à la vente en ligne une portée de sa chienne ou de sa chatte. Toutefois, il supprime la possibilité de proposer sur un site internet la cession à titre gratuit de chiens ou de chats par des éleveurs, donc également par des particuliers détenant la mère. De même, il supprime la cession, à titre gratuit ou onéreux, des nouveaux animaux de compagnie (NAC) par des éleveurs ou des particuliers, puisque la définition d'élevage de l'article L. 214-6-2 se rapporte uniquement aux chiens et aux chats.

source majeure d'abandon et de trafic. Le renforcement des mentions obligatoires et de l'immatriculation des vendeurs ne vont pas assez loin, dès lors que les opérateurs de plateforme ne réalisent pas un contrôle systématique préalable. Avec l'appui des pouvoirs publics, il faut développer des plateformes spécialisées, comportant des règles spécifiques strictes.

Seuls des sites agréés respectant un cahier des charges strict pourront publier de telles annonces, conformes au formalisme légal, renforcé par les dispositions de ce texte, et à la condition que ces opérateurs aient un système de contrôle de la véracité des informations saisies pour mieux lutter contre les trafics.

est à Mme Hélène Conway-Mouret. À l'instar des auteurs de plusieurs amendements qui viennent d'être présentés, nous sommes favorables à l'interdiction de la vente en ligne d'animaux de compagnie sur des plateformes non spécialisées et par des non-professionnels. Nous nous interrogeons, en effet, sur la réelle efficacité du dispositif tel qu'il est proposé aujourd'hui. Il sera très difficile de distinguer les vendeurs professionnels de ceux qui ne le sont pas. Les milliers de petites annonces qui paraissent chaque jour ne pourront jamais être contrôlées, soyons honnêtes ! C'est pourquoi, malgré des avancées rédactionnelles introduites en commission au Sénat, nous considérons que seule une interdiction générale la vente des animaux en ligne sur les plateformes non spécialisées permettra d'obtenir un résultat significatif. Toutefois, nous sommes également sensibles à l'amendement proposé par le Gouvernement, qui nous semble tendre à proposer un bon équilibre.

Le sujet est déjà compliqué techniquement, mais dès que l'on ajoute la dimension internet, il devient compliqué au cube, car l'extraterritorialité nous pose énormément de problèmes. Idéalement, nous

Nous souhaitons préciser que cette interdiction ne concerne que les animaux vertébrés et vivants afin d'exclure notamment les appâts de pêche, les insectes, voire les huîtres ou les crustacés. Il s'agit donc, mes chers collègues, d'un amendement de cohérence.

Ces techniques de marketing favorisent les achats impulsifs et s'inscrivent donc aux antipodes d'une acquisition réfléchie et faite en connaissance de cause d'un animal, lorsqu'il s'agit d'un animal exotique. Il me semble donc que toutes les techniques promotionnelles, quelles qu'elles soient, doivent être bannies : tel est l'objet de cet amendement,

code rural et de la pêche maritime ne prévoit un statut d'éleveur d'animaux de compagnie que pour les éleveurs de chiens et chats. Ce statut s'applique assez largement, puisqu'il recouvre toute personne qui a fait naître d'une femelle reproductrice, puis cédé, au moins un chiot ou chaton. Dès lors, il concerne aussi de nombreux particuliers éleveurs. Il pourrait, dans certains cas, être pertinent d'étudier la création d'un statut d'éleveur pour d'autres animaux, comme le propose M. Bazin : cela pourrait être le cas, par exemple, pour les lapins et les furets. Cependant, l'amendement tend ici à inclure l'ensemble des animaux de compagnie domestiques, ce qui englobe par exemple les canards, les coqs ou les poissons rouges. Je ne suis pas favorable à ce que les Français qui possèdent une mare à canards, un petit poulailler particulier ou un grand aquarium, voire une mare avec des carpes, soient soudainement élevés au rang d'éleveurs professionnels dès lors qu'ils céderaient à un ami l'un des petits

Une poule, un canard, un poisson ne sont pas des animaux de compagnie : je vous renvoie à la réglementation. Un animal de compagnie est un animal que nous détenons pour notre agrément et qui est

L'identification n'est pas obligatoire avant l'âge d'un mois, sauf en cas de sortie du lieu de détention pour les animaux de compagnie non domestiques et, pour les chiens et les chats, en cas de cession avant l'âge respectivement de quatre et sept mois. Tel est l'état de la réglementation. Pourtant, ces animaux peuvent faire l'objet d'une offre de cession à venir

dernier amendement vise aussi à prévoir que la mention du numéro ne sera obligatoire que si les animaux disposent d'un numéro d'identification. La commission n'y est pas favorable, car cela dispenserait tous tous les animaux non identifiés, et ce en dépit des obligations légales. Je rappelle notamment que, au titre de la loi, l'identification des chiens et chats adultes est obligatoire et doit être réalisée à la charge du cédant La rédaction retenue par l'amendement n° 105 rectifié irait à l'encontre de notre objectif, qui est justement d'inciter au respect de la loi. L'avis est donc défavorable.

des frais vétérinaires. Le présent amendement tend donc à compléter les informations figurant sur la publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie en y incluant explicitement une estimation du montant des dépenses nécessaires pour satisfaire les besoins de ces derniers.

du budget consacré aux animaux de compagnie. Je considère que ces propositions, bien qu'intéressantes sur le principe, n'ont pas forcément leur place parmi les mentions obligatoires dans les offres de cession. L'intérêt de ces mentions est plutôt de s'assurer que les offres ne sont pas mensongères et ne cachent pas une fraude. Il appartient par ailleurs à l'acquéreur de se renseigner sur l'ensemble des responsabilités liées à la possession d'un animal de compagnie : les annonces ne peuvent pas se substituer à ses recherches et à la responsabilisation de chacun. Je ne suis donc pas favorable au fait d'alourdir les annonces en y faisant figurer

Pour ne pas avoir à se déclarer, de nombreux annonceurs, vrais ou faux particuliers, proposent des dons ou des cessions à titre gratuit, mais exigent de l'acquéreur, au moment de la remise de l'animal, une contrepartie financière en invoquant une participation aux frais. Le cessionnaire non avisé verse alors généralement plusieurs centaines d'euros au cédant frauduleux. Une étude d'une association, la Fondation Brigitte Bardot, a révélé que 21 % des annonces sont en fait des ventes déguisées en dons. Cette pratique est illégale : elle constitue non seulement une arnaque pour l'acquéreur, mais aussi une concurrence déloyale pour les professionnels qui se conforment aux obligations. Il est donc nécessaire d'interdire clairement cette pratique dans la loi afin que ceux qui acquièrent des chiens et des chats des petites annonces mentionnant un don sachent qu'ils n'ont aucune contrepartie à verser. Quel est l'avis de la commission ?

Cet amendement vise à supprimer les dispositions insérées en commission qui instaurent un système de vérification par les plateformes de la validité des informations contenues dans les annonces en ligne de cession d'animaux de compagnie, au profit du dispositif plus ample et plus ambitieux proposé proposé à l'article 4 . Tout en maintenant cette obligation de vérification par les plateformes, l'amendement que j'ai proposé à l'article 4 vise aussi à instaurer un agrément pour les sites spécialisés de vente d'animaux de compagnie, ainsi que des obligations en matière de sensibilisation et d'information du public.

Les propositions de cession de chiens considérés comme dangereux, dont la loi réglemente la possession, se multiplient. Les annonces en ligne participent également à alimenter les portées effectuées par des particuliers à des fins lucratives, ainsi que le trafic d'animaux transportés dans des conditions lamentables. Il convient donc de responsabiliser les plateformes en instaurant une vérification préalable de la conformité de l'annonce à la loi avant sa publication. nous avons fait un pas significatif, en prévoyant l'obligation pour les plateformes d'annonces de mettre en oeuvre un système de double authentification qui permette de vérifier la fiabilité des informations relatives à l'animal et à son propriétaire, ce dont je me félicite.

Nous avons prévu que les plateformes mettent en oeuvre un système de contrôle préalable suffisant afin de vérifier la validité des informations de l'offre de cession. Pour ces raisons, je demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, j'y serai défavorable.

qui, en dehors de ces sites, publieraient des annonces non conformes. En effet, il me paraît nécessaire d'exercer une forte pression sur les annonceurs eux-mêmes, sur les porteurs de petites annonces autant que sur les sites,

L'article R. 215-5-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit déjà que le non-respect des mentions obligatoires en cas de cession en ligne est puni d'une amende applicable aux contraventions de quatrième classe, c'est-à-dire de 750 euros. Je ne suis pas favorable à l'inscription du montant d'une amende dans la loi, alors qu'elle est déjà fixée réglementairement et, qui plus est, de manière plus dissuasive. J'émets donc un avis défavorable

est l'avis de la commission ? Notre commission n'a pas souhaité introduire de dispositif spécifique aux animaux lorsque des dispositifs de droit commun existent déjà et permettent la même chose. C'est la raison pour laquelle nous avons supprimé le mandat introduit par l'Assemblée nationale, redondant par rapport au droit de la succession et des mandats classiques. L'amendement de notre collègue tend à insérer deux nouveaux articles au sein du code civil, qui prévoient qu'un mandat de protection future peut concerner un animal et qu'un legs peut également porter sur un animal. Je le redis, ces deux propositions sont parfaitement satisfaites par le droit existant. Un décret prévoit ainsi spécifiquement le cas des animaux de compagnie dans les mandats de protection. Il est aussi tout à fait possible de faire bénéficier des fondations et des associations d'un legs d'animal de compagnie. L'inscription du mandataire au fichier national relève du niveau réglementaire. Il ne me paraît pas nécessaire d'alourdir inutilement la loi. J'émets donc un avis défavorable

l'aspect ludique de l'animal de compagnie. L'acquisition d'un animal de compagnie par un mineur n'est pas souhaitable, même avec le consentement parental. Par ailleurs, cet amendement est cohérent article additionnel après l'article 1 qui tend à prévoir qu'un justificatif de domicile validé est nécessaire afin que la détention d'un animal carnivore domestique ne puisse être contestée.

d'un parent, ne me paraît pas aller dans le bon sens. Il arrive souvent qu'un animal acheté pour un jeune de 16 ou 17 ans soit mis à son nom, ce qui contribue à le responsabiliser en tant que maître de l'animal. Je ne souhaite pas interdire

Cette pratique esthétique ancestrale entrave le langage corporel des chiens et leur socialisation. La France est signataire de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie depuis le 18 décembre 1996, dont l'article 10 prévoit que les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites. La réglementation applicable aux interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins curatives serait élevée au niveau législatif, à l'instar des dispositions relatives à l'interdiction de la vente de ces animaux à des mineurs de 16 ans sans le consentement préalable des personnes exerçant l'autorité parentale ou d'autres dispositions de la proposition de loi. Cet amendement vise donc à consacrer dans la loi l'interdiction de la caudectomie.

se trouvent dans cette situation : leurs propriétaires ne paient pas ce qu'ils doivent aux entraîneurs de course ou aux propriétaires de centres équestres.

Afin qu'il remplisse pleinement son rôle, il serait judicieux que cet enseignement soit dispensé par des professionnels du secteur animalier tels que des vétérinaires ou des bénévoles intervenant dans des refuges ou des associations soit axé sur de grandes thématiques : les différentes formes de violences envers les animaux domestiques et sauvages- la sensibilisation serait ainsi double -, la lutte contre l'abandon, etc. Le but est de permettre aux bénéficiaires de ce module de réagir de manière adaptée dans le cas malheureux où ils se trouveraient confrontés à un acte de cruauté envers un animal. Enfin, ils disposeraient ainsi des connaissances nécessaires afin d'accueillir un animal dans leur vie s'ils le souhaitent.

En effet, former les élèves au respect des animaux et à la responsabilité que nous avons envers eux ne pourra que contribuer à la diminution des pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous savons tous que les enfants sont des vecteurs intéressants dans les familles.

au respect de l'environnement et des animaux par un enseignement de l'éthique animale permettrait de prévenir les actes de maltraitance animale chez ces adultes en devenir. Le présent amendement vise à prévoir l'enseignement de l'éthique animale pour les élèves dès le premier et second degrés. L'éducation au développement durable est non pas une matière autonome, mais un enseignement transversal intégré dans toutes les matières. En revanche, l'enseignement moral et civique est évalué lors du brevet des collèges. Il me semble plus pertinent d'intégrer l'enseignement de l'éthique animale à l'enseignement moral et civique.

Il est pour le moins curieux que la chasse à courre et le déterrage soient absents d'un texte qui s'intéresse à tous les sévices que les humains font subir aux animaux dans le cadre de leurs divertissements. Soyons honnêtes : la législation actuelle apparaît comme dépassée et correspond à des pratiques d'un autre temps. Je rappelle que la chasse à courre consiste à poursuivre et à traquer des heures durant, à l'aide d'une meute de chiens, un animal sauvage jusqu'à l'épuisement, la mise à mort étant faite au moyen d'une dague ou d'un pieu.

Il est temps que la France y mette fin, à l'instar de nombreux pays européens- l'Allemagne, la Belgique, l'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles. Si nous ne pouvons pas légiférer sur cette question aujourd'hui, comptez sur nous pour la remettre sur la table jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ces pratiques moyenâgeuses. Il est temps que la France remette en question ce droit acquis à la souffrance animale. Nous venons d'ailleurs de déposer une proposition

Pourtant, il n'est pas de démonstration plus évidente de maltraitance exercée sur des animaux que le spectacle donné dans les arènes mettant en scène la persécution d'un taureau désorienté et sa mort après capitulation, sans étourdissement préalable, Est-il normal que des corridas se déroulent encore en toute impunité dans des régions françaises, au nom de traditions locales, alors que partout ailleurs, sur le territoire français, les actes de cruauté envers les animaux sont sanctionnés d'une peine d'emprisonnement et d'une amende par le code pénal ? La lutte contre la maltraitance animale remet en question l'interprétation d'une loi qui n'est plus réellement adaptée aux attentes de la société et repose encore sur les notions floues de « traditions locales ininterrompues » ou de « courses de taureaux ». Cette législation apparaît désormais comme une tolérance dépassée du législateur et correspond à des pratiques d'un autre temps. Chaque année, au nom de la seule coutume locale, ce sont pas moins de mille taureaux qui sont torturés à mort en France, sans parler de ceux qui meurent lors des entraînements. Pourtant, plusieurs pays qui pratiquaient la corrida ont fait le choix de l'interdire progressivement, comme le Chili, l'Argentine, Cuba ou encore l'Uruguay. La Catalogne a également eu le courage de voter son interdiction en juillet 2010, faisant figure d'exception en Espagne. La France doit elle aussi remettre en question ce droit acquis à la souffrance animale.

de supprimer la dérogation actuelle accordée aux courses de taureaux et aux combats de coqs, car ces animaux appartiennent également à des espèces dont la sensibilité est reconnue par la science.

En ce sens, elle devrait être condamnée au titre de l'article R. 655-1 du code pénal. Or il n'en est rien, le propriétaire pouvant toujours invoquer une nécessité économique ou sociale que les tribunaux lui reconnaissent beaucoup trop facilement. L'euthanasie de convenance est une préoccupation majeure de l'ensemble des associations de protection animale. À cet égard, sa suppression était incluse dans les propositions portées par le collectif AnimalPolitique lors de la dernière élection présidentielle.

Le burn-out compassionnel lié aux euthanasies de convenance a fait l'objet de nombreuses communications scientifiques. Les vétérinaires se sentent coincés par la demande pressante du propriétaire de l'animal et obligés de procéder à un acte qu'ils réprouvent. Enfin, cet amendement appelle par la suite un financement permettant de venir en aide aux animaux susceptibles d'être euthanasiés. Il vise aussi à rendre visible une situation trop souvent cachée.

ainsi à prévoir une réunion collégiale de vétérinaires en cas de demande d'euthanasie non médicalement justifiée. La mise en oeuvre d'une réunion collégiale relève du domaine réglementaire. En outre, on ne voit pas bien ce qu'elle apporterait.

rien n'oblige aujourd'hui les vétérinaires à procéder à une euthanasie qu'ils ne jugeraient pas nécessaire. Tout les pousse, au contraire, à refuser des euthanasies qui ne sont pas médicalement justifiées ; leur conscience, leur expérience et leur professionnalisme demeurent les meilleurs garde-fous contre ces dérives. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

C'est donc un amendement de cohérence que nous défendons, visant à sécuriser un certain nombre d'activités de loisirs ou professionnelles. Quel est l'avis de la commission ?

Quel est l'avis de la commission ? À première vue, il peut paraître surprenant de prévoir une exonération de peine pour les élus et les responsables syndicaux. Au nom de quoi seraient-ils irresponsables de leurs actes de maltraitance commis sur des animaux ?

toute personne peut déjà être exonérée de responsabilité pénale pour un délit qu'elle aurait commis afin de sauver une personne ou un bien. Or, de jurisprudence constante, les

je partage la crainte de l'auteur de l'amendement de voir des personnes se dédouaner de leur responsabilité et tenter d'échapper à cette circonstance aggravante en arguant de de leur inconscience ou de leur négligence. On est en droit d'attendre du propriétaire ou du détenteur d'un animal qu'il soit conscient des situations qui peuvent présenter un risque de mort pour ce dernier. Sinon, ce serait le signe que le certificat d'engagement et de connaissance prévu à l'article 1 ne fonctionne pas. En conséquence, monsieur le ministre,

Quel est l'avis de la commission ? Ainsi, un propriétaire qui abandonnerait son animal, mais qui par ailleurs se soucierait de son sort ou chercherait à s'en occuper, ne serait pas coupable d'abandon. Ce serait lui donner un moyen facile de se dédouaner en lui permettant d'arguer que, pris de remords, il a tenté de retrouver son animal quelques jours après l'avoir abandonné. Laissons plutôt le juge

En France, environ 1 300 chiens travaillent aux côtés de nos policiers et de nos gendarmes. Ils font partie intégrante de nos effectifs de police et de gendarmerie. Ces chiens participent aux opérations de police préventives et répressives, en cas de menace réelle et sérieuse. Lors de leurs différentes interventions, les chiens policiers font souvent l'objet d'attaques. Ils sont ainsi maltraités, brutalisés, frappés lors de contrôles et d'interpellations, sans que les coupables ne puissent être véritablement inquiétés.

l'avis du Gouvernement ?

Ces limites permettent donc aux prévenus de tricher et de garder l'animal en prétendant ne pas en être le propriétaire. Par exemple, les fiches d'immatriculation peuvent ne mentionner qu'un seul propriétaire, ce qui permet aux prévenus d'immatriculer l'animal au nom de leur conjoint et ainsi d'éviter toute confiscation. Il nous a paru

des responsabilités syndicales. Cette peine complémentaire prévoit l'interdiction de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale, dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.

Quel est l'avis de la commission ?

de céder ou de faire adopter plus facilement un animal retiré à son propriétaire, mis en cause pour maltraitance animale, dans l'attente de son jugement. Il tend ainsi à apporter une solution au problème de la saturation des refuges, qui est due à la lenteur des procédures judiciaires. Pour autant, le présent amendement a pour objet de supprimer le nouveau critère de prise en considération « des besoins physiologiques propres » à l'espèce,

les directions départementales de la protection des populations (DDPP). Ces acteurs de terrain sont aujourd'hui contraints de refuser les retraits d'animaux par manque de place, ce qui conduit à des situations dramatiques. dramatiques. La procédure de cession avant jugement, prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, respecte la présomption d'innocence et le droit de propriété car, si le propriétaire mis en cause pour maltraitance est relaxé, le produit de la vente lui est intégralement reversé. Les associations de protection animale nous expliquent d'ailleurs que, quand un propriétaire tient réellement à son animal, il le leur réclame et qu'elles le leur rendent bien volontiers quand il semble être de bonne volonté.

pas. En cas de confiscation, en effet, l'animal est confié à une association de protection animale. En aucun cas, l'ancien propriétaire ne peut se retrouver en sa détention. Il n'y a donc aucun problème de bonne application de la peine dans cette

Les chiens utilisés par les agents cynophiles sont parmi ceux que l'on retrouve en majorité en fourrière et en refuge. Les associations de protection animale sont régulièrement appelées à la suite de la découverte de chiens d'agents cynophiles maltraités. Ces chiens sont détenus en dehors ou non des horaires de travail dans des conditions particulièrement indignes et enfermés en continu

Il est donc souhaitable que, au même titre que les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d'animaux, ces agents cynophiles, comme leurs employeurs, puissent être sanctionnés par une infraction délictuelle, tel que le prévoit et le réprime l'article L. 215-11 du code rural Il convient également de préciser que l'on constate régulièrement que ces chiens servent indifféremment à différents agents cynophiles non déclarés auxquels ils sont prêtés sans que, pour autant, ceux-ci en soient les détenteurs inscrits au fichier national

Je remercie mon collègue Arnaud Bazin de proposer d'inclure les entreprises d'agents cynophiles dans la liste des professions exerçant en lien avec les animaux, au même titre que les entreprises de toiletteurs ou d'éleveurs aujourd'hui. Elles pourront désormais encourir les peines pour mauvais traitements prévues à l'article L. 215-11

pour ne pas avoir su prévenir de telles dérives. Les sanctions prévues par ledit code s'appliquent aux établissements professionnels. Pour les particuliers, il y a le code pénal. Il serait curieux et légèrement discriminatoire que les agents cynophiles soient les seuls salariés visés ; ce n'est en effet le cas d'aucune autre profession.

par la jurisprudence : elle définit un contact à caractère sexuel avec un être vivant qui ne peut pas exprimer son consentement. Si les termes « atteintes sexuelles » s'appliquent uniquement aux mineurs, il n'y a bien sûr aucune assimilation entre animaux et enfants. D'ailleurs, les peines montrent bien qu'il ne s'agit pas de la même chose : les atteintes sexuelles sur mineur sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende,

elle constitue évidemment une déviance qui s'accompagne, dans la moitié des cas, de sadisme. Les sites spécialisés sont aisément accessibles, y compris par les mineurs, et recevraient environ 1,6 million de visites chaque mois en France selon l'association Animal Cross. La consommation des images crée l'offre. Or les condamnations pour sévices de nature sexuelle sur animaux sont rares et la répression des atteintes sexuelles sur les animaux constitue une réponse insuffisante. Le présent amendement a pour objet de rétablir la sanction applicable en cas de consultation habituelle de zoopornographie

habituelle de sites terroristes et de sites pédopornographiques tombe aujourd'hui sous le coup de la loi. Le Conseil constitutionnel est très attentif à la proportionnalité et avait censuré une première fois le délit de consultation habituelle de sites terroristes. Nous renforçons les sanctions pour sévices sur animaux et créons un délit d'atteinte sexuelle. Ce sont déjà des avancées majeures.

Les comportements zoophiliques, jusqu'à l'invention d'internet, étaient marginaux, peu visibles. Ils posaient assez peu de problèmes à la société parce qu'ils ne concernaient vraisemblablement

Comment un vétérinaire peut-il savoir que l'auteur des coups a agi en vue de faire souffrir, c'est-à-dire caractériser le caractère intentionnel de l'acte ? Les vétérinaires devraient constater eux-mêmes ce qui relève ou non d'un délit avant de pouvoir lever le secret professionnel. leur appartient pourtant pas de constater l'existence d'un délit. Ils ne peuvent que constater des manifestations cliniques ou comportementales pouvant laisser penser à un acte de maltraitance répréhensible pénalement. C'est du reste ce que précise le code de déontologie vétérinaire.

En plus de sanctionner les personnes qui proposent, sollicitent ou acceptent des petites annonces zoophiles, le dispositif prévoit de réprimer ceux qui incitent à la commission de l'un des faits visés au futur article 521-1-1 du code pénal.

Pour sanctionner ces sites, il convient de punir toute entité qui aurait permis de commettre l'une des infractions prévues à l'article 521-1-3 du code pénal. Sans ces sites, il est supposé que la commission de l'une de ces infractions n'aurait pas été possible : le site internet met à disposition les moyens nécessaires pouvant conduire à la commission des infractions.

La zoophilie constituant également une déviance sexuelle, son inscription au Fijais peut servir à prévenir certaines dérives. Cette inscription permettrait à terme d'élaborer un fichier des personnes condamnées ou poursuivies pour des infractions envers des animaux. Il existe un lien bien établi entre les agressions sexuelles sur les animaux et les agressions sexuelles sur les êtres humains. Le sujet a été étudié par plusieurs criminologues aux États-Unis. Selon une étude de Jenny Edwards publiée en 2019, 32 % des personnes arrêtées pour des actes de zoophilie aux États-Unis avaient aussi agressé sexuellement des enfants et des adultes ; 53 % d'entre elles avaient un dossier judiciaire avec des agressions sexuelles sur des êtres humains, des actes de violence, des délits liés à la drogue ou des atteintes aux biens. Selon deux autres études, 38 % de prisonniers masculins incarcérés pour des agressions sur des enfants ont aussi agressé sexuellement des animaux

monsieur le ministre, soit proportionnée et pertinente. Il en va ainsi de l'inscription au fameux Fijais. Les infractions susceptibles d'entraîner une inscription dans ce fichier sont parmi les plus graves sur l'échelle des valeurs sociales. Placer au même niveau les actes sexuels et les violences sur les personnes et les infractions-

Bouglione. « Le cirque animalier, dit-elle, peut paraître un sujet mineur, comparé à tout ce que subissent par ailleurs les animaux. Néanmoins nous exerçons une certaine influence sur les mentalités et sur le regard que la société porte sur les animaux, dès la plus tendre enfance de notre public, de génération en génération. « Heureusement, les temps changent et la société évolue. Aujourd'hui, l'idée de maintenir en captivité des animaux sauvages appartenant à des espèces en voie d'extinction dans leur milieu naturel, dans l'unique but de les exhiber dans des spectacles à destination des familles, et plus particulièrement des enfants, est devenue insupportable pour la grande majorité de la population. Ils sont merveilleusement beaux et charismatiques, et comme tout le monde veut les voir en vrai, nous nous permettions de les emprisonner à vie, eux et leur descendance. Ils sont donc victimes de leur beauté et de leur charisme, que l'on donnait à " consommer " le dimanche, en famille. Ce fut donc pour nous mettre en accord avec nous-mêmes, et aussi pour tenir enfin compte de l'évolution positive de la société sur la question animale, que nous avons finalement décidé de ne plus jamais exploiter d'animaux dans nos futurs spectacles. Dans le monde de l'exploitation animale, le cirque animalier occupe une place importante. Il convient de l'arrêter en premier, car [cette exploitation] est non seulement la plus futile et la plus inutile, elle est aussi celle qui a le plus de conséquences néfastes sur notre perception erronée du statut des animaux dans notre société. »

ayant conduit la commission à proposer une solution de compromis. Pour les spectacles itinérants, il s'agit d'une liste mentionnant l'ensemble des animaux non domestiques dont la détention est interdite pour ces spectacles, liste établie après une concertation générale avec l'ensemble des parties prenantes, professionnels et experts. Le rythme d'interdiction est adapté selon le degré d'adéquation des besoins physiologiques de l'animal avec le mode de vie itinérant. Cette solution n'est pas originale. Elle recoupe en grande partie, en l'enrichissant, la version initiale de la proposition de loi. Je rejoins donc les rapporteurs de l'Assemblée nationale dans leurs travaux initiaux et ceux qui prétendent que le Sénat dénature le texte se trompent. Nous revenons à son essence, en débattant de modalités d'application de l'article respectueuses des professionnels, ce qui, à terme, mes chers collègues, vous aidera à prendre une décision fondée.

Le risque lié à une interdiction sans concertation et sans consensus est de créer des effets de bord. Les professionnels des parcs aquatiques sont, par exemple, à l'origine d'avancées en matière de recherche sur l'éthologie des dauphins, permettant de mieux comprendre, aussi, les comportements de ces animaux en mer.

non cancérogène ne trouvent pas de solution et de réponse dans l'immédiat. Il me paraît donc extrêmement difficile de vous donner gain de cause sur ce sujet. Voilà ! Le décor est planté

d'instaurer une interdiction, pour les établissements itinérants détenant des animaux non domestiques et pour les établissements détenant des cétacés. d'une nouvelle rédaction de l'article 12, est revenu sur l'interdiction générale pour les cirques détenant des animaux non domestiques, ainsi que pour les montreurs d'ours et de loups, de commercialisation, transport, acquisition, reproduction des animaux et ouverture de nouveaux établissements. Cette nouvelle rédaction prévoit également de nombreuses dérogations. Mes chers collègues, de plus en plus de communes refusent d'accueillir des cirques détenant des animaux ; de plus en plus de nos concitoyens se détournent du spectacle d'animaux sauvages, trop souvent malheureux. Quel animal sauvage passant sa vie enfermé dans une cage, transporté, privé d'espace et de liberté et exposé sur une piste ou ailleurs, à réaliser des numéros devant une foule bruyante, peut en effet se sentir bien ? Nous pouvons entendre la nostalgie, celle des spectateurs et des circassiens qui voient leur mode de vie et de représentation changer, mais il est temps que ces pratiques s'éteignent et que nous proposions à nos enfants une autre vision que celle de malheureuses bêtes exposées sous les lumières et enfermées dans l'ombre. Les arts magnifiques du cirque se diversifient et continuent de nous faire rêver, nous et nos enfants. Ils peuvent le faire sans maltraiter d'animaux. Au spectacle sordide de l'enfermement, nous préférons le respect du vivant, ainsi que la diversité et la créativité que le cirque est capable d'offrir. C'est pourquoi nous proposons de rétablir l'article 12 dans sa version initiale, telle qu'elle a été proposée et votée par l'Assemblée nationale.

excepté les établissements zoologiques, et pour l'ensemble des animaux d'espèces non domestiques dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. L'itinérance est un facteur aggravant, mais les problèmes majeurs sont bien le dressage et la captivité, sans parler du risque lié à la sédentarisation des cirques itinérants ou du cas des montreurs d'ours. Nous déplorons, madame la rapporteure, le recul de la commission par rapport au texte initial. La rédaction de la commission prévoit de nombreuses dérogations et ne répond donc aucunement à la volonté des Françaises et des Français, dans leur immense majorité, d'en terminer avec la détention et l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums et autres établissements de spectacle.

est déjà en vigueur dans 23 des 27 pays de l'Union européenne -et 69 % se déclarent favorables à l'interdiction des delphinariums. Mais le plus important, c'est que le bien-être des animaux détenus et utilisés par les établissements de présentation publique ne peut pas être assuré en raison de multiples déplacements, de la limitation et de l'inadéquation de l'espace disponible, ainsi que de la contrainte exercée pour réaliser des mouvements et des prestations inadéquates. la Fédération des vétérinaires d'Europe a ainsi recommandé à toutes les autorités compétentes, européennes et nationales, d'interdire l'utilisation de mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute l'Europe, compte tenu de l'impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux. Quel